Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec une très grande émotion qu'une attaque s'est produite, ce matin, dans le périmètre de la basilique Notre-Dame de Nice. D'après les informations dont nous disposons à cette heure, plusieurs personnes auraient été tuées et d'autres blessées. Dans ces circonstances tragiques, nos pensées vont bien sûr aux victimes et à leurs familles : ce qui vient de se passer nous bouleverse tous.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

Les opérateurs se retrouvent alors sans aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet, qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières.

Cet assouplissement se justifie d'autant plus que de nombreux laboratoires de recherche travaillent sous tutelles communes- EPST, EPIC et fondations. Les facilités proposées seront toutefois encadrées : un décret en Conseil d'État fixera la nature des chantiers ou opérations de recherche pour ce type de contrat, les modalités de recrutement, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié, et les mesures d'accompagnement de ce dernier une fois le contrat achevé. En outre, il est proposé que le décret fixe un quota maximal de CDI de chantier par rapport à l'effectif global de l'établissement. Ce quota pourrait s'établir autour de 10 %. Quel est l'avis de la commission

L'article 6 s'inscrit dans l'objectif de revalorisation des métiers de la recherche visé par le présent projet de loi. Il tend à lutter contre la précarité des doctorants et jeunes chercheurs titulaires d'un doctorat, qui assurent souvent des heures d'enseignement sous la forme de vacation lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un contrat, en garantissant le paiement mensuel de ces heures d'enseignement. Le présent amendement a pour objet d'avancer l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1 septembre 2021, au lieu du 1 janvier 2023.

est à M. Christian Redon-Sarrazy. L'article 6 a été fort heureusement introduit lors du débat en séance à l'Assemblée nationale. Ce dispositif devrait permettre de mettre fin aux retards de paiement des vacataires, qui accentuent encore un peu plus le caractère précaire de leur statut.

J'en profite pour m'interroger sur l'adéquation du dispositif, qui, en complétant l'article L. 952-1 du code de l'éducation, vise les conditions d'emploi des seuls chargés d'enseignement, et non celles des agents temporaires.

l'avis du Gouvernement ? Comme vous l'avez rappelé, madame la rapporteure, je suis extrêmement favorable à ce que nous puissions régler, une fois pour toutes, le problème du paiement des vacataires.

Il faut bien comprendre la situation dans laquelle se trouvent à la fois les contractuels et les universités. Aujourd'hui, les universités- je les ai consultées -expliquent être dans l'incapacité d'appliquer la disposition que nous allons voter,

plus vaste, pour tenter de comprendre comment un certain nombre de missions de service public sont assurées, à l'heure actuelle, par des moyens aussi peu conformes aux règles de la fonction publique. Je

celui-ci a été réduit à trois ans en 2010, voire à deux ans, compte tenu du maintien en activité en surnombre d'un an dont certains professeurs peuvent bénéficier. de ce différentiel de cinq ans, au moins, avec les professeurs des universités permettra de prendre de nouveau en compte les spécificités des missions du Collège de France.

disposition concerne un nombre très limité d'enseignants- moins de 50 -, les plus éminents dans leur spécialité, dont l'aura est internationale. En plus d'une recherche de haut niveau, ces derniers assurent, depuis 1530, la diffusion de la culture scientifique auprès d'un large public, récemment par le biais de podcasts très populaires.

qu'ils bénéficient, ou non, d'un recul de limite d'âge pour motif familial. Ce surnombre permet aux professeurs d'être maintenus en activité après la limite d'âge et de continuer à acquérir des droits à pension. Le présent amendement du Gouvernement vise à rétablir une durée homogène d'un an de surnombre pour tous les professeurs de l'enseignement supérieur : il est prévu que ce surnombre prendra effet à la limite d'âge ou à l'issue d'éventuels reculs de limite d'âge.

d'un amendement en commission a fait passer cet âge limite à 70 ans, alignant ainsi toute carrière de professeur sur celle des professeurs du Collège de France, et ce sans motif justifiant ce recul d'âge de départ. Par ailleurs, le présent projet de loi prolonge potentiellement de cinq ans la carrière des professeurs responsables d'un projet lauréat. Ceux-ci pourraient ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'à l'âge de 72 ans. On s'interrogera sur la notion même d'équipe portant un tel projet et sur la nécessité d'une transmission et d'une passation de pouvoir à un autre membre de l'équipe, lesquelles ne nécessitent assurément pas une durée de cinq ans pour qui est déjà associé à des travaux ! Notre amendement tend ainsi à reculer au maximum d'un an la date de départ à la retraite, indépendamment du motif de retard de ce départ.

au lauréat d'un appel à projets puissent continuer à être versés, même dans le cas où celui-ci aurait atteint cette limite. Il s'agit d'un cas très circonscrit, qui doit seulement permettre que la conduite des projets concernés ne soit pas remise en cause. L'avis de la commission est

la procédure d'autorisation à rester en fonction au-delà de la limite d'âge pour continuer d'exercer la responsabilité d'un projet lauréat d'un appel à projets, à l'instar de la procédure d'attribution de l'éméritat. est l'avis de la commission ? Cette procédure de maintien en fonction étant exceptionnelle, elle doit être autorisée par un acte réglementaire de niveau ministériel, et non par un simple avis d'une commission interne à l'université. L'avis de la commission est

est à Mme la ministre. L'élaboration de la stratégie nationale de recherche en 2014 a permis une consultation large et une expression claire des grands enjeux, grands enjeux, mais sans dégager de réelles priorités nationales qui puissent se traduire dans une programmation opérationnelle. De façon récurrente, dans le champ de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, une stratégie nationale aboutit très souvent à un texte dans lequel chaque discipline et chaque thème est évoqué sans réelle différenciation. Il s'agit donc de remplacer l'objet que constitue la « stratégie nationale de la recherche » par des orientations prioritaires de la politique nationale de recherche, qui seraient mises en oeuvre par contractualisation avec les établissements, déploiement de programmes prioritaires de recherche ou programmations de l'Agence nationale de la recherche,

le ministre, six scientifiques, un député, un sénateur et un représentant de Régions de France. L'amendement

Avec l'amendement n° 231, le Gouvernement propose une réforme structurante de la stratégie nationale de recherche, laquelle n'a pas eu, jusqu'à présent, les effets escomptés. Le ministre ne se contenterait pas de coordonner cette stratégie : il arrêterait des orientations prioritaires après une large consultation des acteurs concernés.

défaut majeur de votre gouvernement : vous ne prenez jamais le temps de consulter la représentation nationale et d'agir dans le cadre des lois. Vous préférez systématiquement réunir des commissions,

La pandémie de la covid-19 constitue un véritable paradoxe pour le débat scientifique. Certes, ce dernier se trouve placé sous le feu des projecteurs et permet de sensibiliser avec acuité les citoyens aux questions scientifiques. Mais il n'échappe pas à ces écueils de la médiatisation en continu que sont le débat de postures, l'invective et la réaction à chaud. Ce format sied particulièrement mal au débat scientifique, qui- on l'a dit -se nourrit du temps long, de la réflexion, des expérimentations menées et de ses conclusions empiriques. L'ampleur de l'enjeu politique, économique et sociétal que représentent la lutte contre le coronavirus et son corollaire- la découverte d'un vaccin -a également accentué cette tension, cette pression du résultat conduisant à l'affirmation de faits qui n'étaient parfois, en réalité, que des hypothèses. En ce sens, le déplacement du débat scientifique d'un espace traditionnellement littéraire, par articles et revues interposés, à un espace plus médiatique a substitué au régime de l'hypothèse et de la preuve scientifiques celui de la vérité autoritaire, mais non moins spécieuse. En d'autres termes, la logique même de la science a été perdue de vue par instants. On constate ainsi l'impérieuse nécessité de renforcer l'intégrité scientifique. Cette problématique- précisons-le d'emblée -ne vise à restreindre ni la liberté d'expression ni les libertés académiques des chercheurs et des enseignants. La science a toujours progressé grâce aux polémiques et aux controverses. Dans une large mesure, elle est même un art de la controverse. C'est d'ailleurs pourquoi les arguments d'autorité sont si peu pertinents dans le champ scientifique. Néanmoins, le pendant de ces libertés réside précisément dans l'intégrité scientifique, qui est une forme d'exigence à l'égard du monde de la recherche. En faisant appel aux notions d'impartialité et d'objectivation de la connaissance, cette intégrité participe de ce qu'on pourrait appeler une éthique scientifique. Sans elle, nous basculons de la connaissance vers l'opinion, de la recherche de la vérité vers la clameur du fait erroné. Or la science n'est pas déconnectée de la société. Au contraire, dans cette période délicate, par tant de soubresauts, elle est un repère et un espoir pour nombre de personnes. Mais elle se doit de conserver sa rigueur, caution de sa crédibilité, faute de quoi- on le sait -la confiance que leur portent les citoyens s'érodera ; et alors, elle se verra attaquer plus avant, comme l'ont été toutes les institutions, par la suspicion, la défiance et la post-vérité ! La parole

notre rapport dans une quinzaine de jours. Aujourd'hui, la France, comme d'autres pays dans le monde, est victime de méconduites scientifiques. Ces dernières

Premier ministre, M. Castex : « Nous assumons qu'il faut que les chercheurs publient, qu'ils aient des résultats à l'appui des moyens que l'on met. Nous allons mettre beaucoup de moyens dans la recherche, il faut que notre production s'en trouve améliorée. »

ouverte. En réalité, rien ne révèle mieux la qualité d'un article que la capacité qu'ont les pairs de s'en saisir. L'amendement n° 100, présenté par MM. Ouzoulias

elles développent ainsi des procédures et des modalités qui leur sont propres. Ces dispositions sont adaptées à la spécificité des écoles de commerce et d'ingénieurs, lesquelles ont bien sûr pour mission de former des ingénieurs et des cadres aux compétences adaptées aux besoins des entreprises françaises.

L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est à Mme la ministre. Il s'agit, par cet amendement, de préciser dans la loi la procédure de désignation du président du Hcéres, avec un appel public à candidatures et un examen des candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre. La mise en place de cette procédure me semble répondre à une obligation de transparence, même si les textes ne l'imposaient pas. C'est d'ailleurs ainsi que cela a été fait en 2020. Les autres modifications proposées sont rédactionnelles.

Le collège du Hcéres est vacant depuis un an. La semaine passée, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a auditionné M. Thierry Coulhon pour se prononcer sur sa nomination en tant que président,

Toute la procédure de sa candidature a été entachée d'un manque total de sérieux et de transparence. Afin d'éviter qu'un tel scandale ne se reproduise, nous proposons de consacrer la qualité

l'amendement n° 101, le principe du contradictoire, qui permet aux évalués de faire connaître leur point de vue sur leur évaluation, est une condition de la légitimité et de l'acceptabilité de celle-ci ; l'avis de

concernées redoutent en effet une perte d'indépendance de la CTI et de la CEFDG dans la définition de leurs référentiels, qui sont reconnus à l'international. Dans la pratique, il existe bien une harmonisation et une coordination des procédures d'évaluation

Cet amendement vise donc à élever au niveau législatif la procédure mise en place lors de la dernière nomination du président, soit un appel public à candidatures et un examen de ces candidatures par une commission. Cette initiative semble apporter toutes les garanties, puisqu'elle sera complétée par l'examen rigoureux mené par les commissions au titre de l'article 13 de la Constitution. Nous émettons donc un avis favorable et j'ai le sentiment de me faire le porte-parole de l'ensemble de mes collègues en indiquant qu'il aurait été bienvenu qu'une telle évolution

Par ailleurs, l'usage systématique de l'anglais recouvre une réalité économique qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, les revues qui publient l'essentiel des travaux scientifiques sont anglo-saxonnes

et des publications scientifiques dans des revues anglo-saxonnes, nous essayons d'ajouter un peu de diversité et de permettre à la France de regagner sa souveraineté scientifique, qu'elle a perdue au profit

que nous devons baisser pavillon. Notre très belle langue a une richesse et une finesse que n'a pas la langue anglaise. Comme l'écrit Pierre Ouzoulias dans l'exposé des motifs, le fait de pouvoir publier en langue française permet d'exprimer avec encore plus d'acuité certains faits scientifiques. Bravo, donc, pour cet amendement, que nous serons très nombreux à soutenir.

sur la manière dont une forme d'uniformisation culturelle s'impose, par facilité et par renoncement. Je demande aux autorités françaises

J'ai demandé au secrétariat général du Sénat de m'indiquer combien de chercheurs du CNRS ou des universités venaient déposer devant les commissions sénatoriales, apportant leurs compétences et leur expertise.

Alors que la crise sanitaire a révélé l'importance, mais aussi toute la difficulté de l'expertise scientifique, il importe de valoriser les actions des chercheurs en direction de la sphère publique. Nous en avons souvent parlé au sein de l'Opecst ; l'avis de la

loi, les évaluations se font sur l'ensemble des missions et des objectifs fixés par le code de la recherche et le code de l'éducation ; l'apport d'expertise en appui aux pouvoirs publics en fait partie.

de connaître les résultats dans le domaine de la publication scientifique des efforts considérables consentis par la Nation par le biais de ce

l'avis de la commission ? l'avis du Gouvernement ?

À travers cette politique, il s'agirait notamment de rendre plus accessibles les médicaments en termes de coût et plus transparente la traçabilité des innovations financées sur fonds publics.

quant à l'esprit général- d'un point de vue fonctionnel, c'est un peu plus compliqué. Madame la ministre, j'aimerais que vous vous engagiez en séance sur la capacité de l'Office français pour l'intégrité scientifique à mener une politique parfaitement indépendante de celle du

Ce nouveau cadre doit permettre aux établissements de se doter d'un corpus de prescriptions en matière d'intégrité scientifique, afin d'outiller davantage leurs référents et, ce faisant, de garantir l'honnêteté et la rigueur scientifique des travaux de recherche menés en leur sein.

l'avis du Gouvernement ?

qui ajuste les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 en associant les collectivités territoriales aux contrats conclus entre les sites universitaires et l'État. de préciser que le volet territorial des contrats de site est élaboré au regard des objectifs et des moyens envisagés, à partir d'une étude d'impact qui lui est annexée ; celle-ci porte sur les effets locaux et régionaux de développement durable et culturel du site universitaire et de recherche. Cette étude d'impact vise notamment à mesurer les évolutions et les risques auxquels sont confrontés les services publics de la recherche et de l'enseignement supérieur sur le territoire considéré. Elle doit permettre d'accompagner et de protéger les petites villes pourvues de sites déconcentrés.

mettent en évidence la nécessité de développer des évaluations partenariales et de sensibiliser les associations d'élus à cette problématique ». Conformément à l'esprit de la loi de 2013 et aux schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui en sont la traduction, notre amendement sert les objectifs de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur dans les territoires ruraux, d'aménagement du territoire par l'activité de recherche et, plus généralement, de réduction des inégalités territoriales.

me semble très prometteur. En revanche, je suis réservée sur votre amendement, dont l'adoption imposerait de réaliser une étude d'impact avant même d'avoir commencé à mettre en place l'association des collectivités territoriales aux contrats des sites universitaires.

à inscrire les modalités de gouvernance, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet dans le code de la recherche, tout en clarifiant ses compétences en matière de coopération scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. à inscrire ce campus dans son territoire, en prévoyant un volet spécifique du contrat d'établissement associant les collectivités territoriales, notamment la région d'Île-de-France.

Mon cher collègue, la prestation de serment que vous proposez n'a pas valeur seulement de symbole. Elle participe aussi à la nécessité de mieux valoriser le doctorat et de sensibiliser le jeune docteur aux principes d'honnêteté et de rigueur qui sont au fondement de l'intégrité scientifique. Avis favorable. l'avis du Gouvernement ?

actuelle, l'article 11 aggrave la complexification du paysage de la recherche publique française, puisqu'il permet la création directe d'unités de recherche par d'autres établissements, sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

La logique d'uniformisation est bien sûr tout à fait louable, mais elle est en totale contradiction avec le principe d'autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent

sénateur, la limitation que vous proposez constituerait un problème fondamental pour certaines associations et fondations, qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs de la recherche publique, comme l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie,

que parce qu'elles sont installées, reconnues et financées par un ou plusieurs opérateurs ; elles fonctionnent évidemment dans le cadre d'une politique globale définie par leur tutelle. La confiance que nous

L'une des principales craintes exprimées par le monde de la recherche concernant le présent projet de loi de programmation est en effet qu'il ne conduise à accentuer la concentration des crédits au profit des plus gros pôles de recherche. Madame la ministre, nous le comprenons bien, c'est justement pour éviter cet écueil que vous avez choisi de faire transiter l'augmentation des crédits par l'Agence nationale de la recherche. Il est clair qu'un financement direct des laboratoires conduirait mécaniquement à accentuer les inégalités territoriales, car les laboratoires seraient alors financés en fonction des budgets des universités, qui eux-mêmes sont historiquement construits, et donc peu équitables. En revanche, il n'est pas certain que l'Agence nationale de la recherche permette mécaniquement d'éviter l'écueil de la concentration des crédits, tout simplement parce que les plus gros pôles de recherche sont aussi les mieux équipés pour répondre aux appels d'offres. Les élus locaux que nous sommes savent bien qu'une collectivité plus importante que d'autres dispose de ressources en ingénierie également plus importantes ; ce sera la même chose pour les laboratoires. Pour éviter l'accentuation de la concentration des crédits liée à la mécanique de l'Agence nationale de la recherche, le présent amendement vise donc à lui imposer de les répartir en prenant en compte un certain équilibre territorial. L'intention est louable, cher collègue, mais ne semble guère compatible avec le principe de sélection des projets de recherche sur la base de critères avant tout scientifiques. La prise en compte d'un critère de répartition territoriale entraînerait une complexification du système qui n'est pas souhaitable. Je demande le retrait de cet amendement.

et de l'innovation sur la répartition du préciput « nouvelle formule », ce que la commission appelait de ses voeux. Lors de son audition, la ministre nous a annoncé quels seraient les bénéficiaires- les établissements gestionnaires, les établissements hébergeurs, les laboratoires et les politiques de site -et à quelle hauteur. Toutefois, nous ne retrouvons absolument pas ces éléments dans l'amendement

sur l'amendement n° 131 rectifié

autonomes et responsables, à décider des règles communes de répartition de ce préciput dans le cadre de leur politique scientifique partagée. Il me paraît que la solution la plus appropriée consiste à inclure les dispositions correspondantes dans les accords de recherche conclus entre établissements. établissements. En l'absence de consensus, un décret peut fixer des règles de répartition, sans perdre de vue l'objectif de financement visé au travers de cet amendement, notamment sur la stratégie de recherche. Nous devons encourager la collaboration entre établissements de recherche, car elle fait la richesse du système français. À cette fin, il est nécessaire, pour prendre en compte les frais indirects des projets de recherche, notamment liés à l'environnement et à la gestion, et accélérer leur conduite, de préconiser des pratiques contractuelles de répartition de ces coûts entre les différents établissements.

et financer des projets qu'ils voient émerger sans qu'il leur soit nécessaire de demander des financements spécifiques à leurs établissements de tutelle. Il ne s'agit pas de centaines de milliers d'euros ; il s'agit de pouvoir leur donner

Monsieur Ouzoulias,

une vache à lait, si je puis dire, pour un certain nombre de politiques publiques que vous pourriez parfaitement soutenir par un autre mode de financement, notamment par la distribution des crédits récurrents.

à des projets en sciences humaines et sociales. Il faut sortir de l'idée que les sciences humaines et sociales dans notre pays ne sont pas capables de

La qualification d'Eespig nécessite que les formations et les diplômes visés ou conférant grade soient adossés à la recherche, ce qui impose qu'on puisse reconnaître une activité de recherche à ces établissements. Vous souhaitez qu'un dialogue financier soit prévu tous les trois ans. ans. L'élaboration du contrat pluriannuel d'établissement entre l'État et les Eespig comprend déjà une annexe financière et permet donc ce dialogue régulier. Enfin, vous souhaitez l'introduction d'un nouveau chapitre dans le code de la recherche comprenant un article unique relatif aux Eespig

la prochaine séance. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Pierre Jourdan, qui fut sénateur de l'Ardèche de 1971 à 1980. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières est parvenue à l'adoption d'un texte commun.